qui leur demande de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés. Ces difficultés sont liées au manque d’outils pour mesurer les inégalités sociales à l’école ; mais elles sont aussi dues à l’attitude de certains établissements privés et au chantage à la fermeture que plusieurs d’entre eux exercent pour obtenir des subventions complémentaires.

certains parmi vous pensent qu’il faut sortir des caricatures et que l’enseignement privé prend déjà toute sa part pour répondre à l’impératif de mixité. Pourtant, le rapport de juin 2023 de la Cour des comptes établit sans appel que « la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat est en fort recul depuis une vingtaine d’années ».

Je m’indigne que le désinvestissement de l’État dans l’école publique pousse de plus en plus de parents à inscrire leurs enfants à l’école privée ; et je m’indigne que les collectivités soient laissées seules face à cette situation. La liberté de l’enseignement n’est pas remise en cause par ce texte. Elle est d’ailleurs protégée par la décision du Conseil constitutionnel de 1977. Ce que nous demandons, c’est qu’elle s’exerce en toute équité et que les écoles privées ne soient pas avantagées au détriment des écoles publiques. Charité bien ordonnée commence par soi même.

tendent à concentrer les élèves de milieux favorisés, ceux qui bénéficient d’un encadrement familial plus fort et qui ont hérité d’un capital culturel plus important, qui peuvent ainsi réussir plus aisément à niveau d’effort égal, tandis que d’autres écoles, publiques ou privées également, suivent le chemin inverse et concentrent les difficultés. La publication des indices de position sociale met en lumière de manière indiscutable et précise la réalité des inégalités socioscolaires sur l’ensemble du territoire national. Les IPS sont des outils

le partage de l’excellence, pour que chaque enfant, quel que soit son milieu, puisse s’épanouir et développer son plein potentiel. C’est cette société juste et équitable que nous devons défendre, car elle permet de mesurer notre capacité d’offrir à tous les enfants

chers collègues, en votant cette proposition de loi, nous ne faisons pas qu’un choix politique, nous réaffirmons toutes et tous notre engagement envers les valeurs et les principes fondamentaux de la République. Si nous aspirons collectivement à former des citoyens éclairés, capables de contribuer pleinement à la vie démocratique de notre pays,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

fragilisée et fracturée à l’image de la France d’aujourd’hui. Les indices de position sociale attestent la persistance de très importants écarts dans la composition des écoles, collèges et lycées. L’école devrait logiquement refléter la diversité de la population française et réunir des jeunes d’origines sociales, géographiques et culturelles différentes. En leur permettant d’apprendre et de grandir ensemble, elle a vocation à être le creuset de la cohésion nationale. C’est pourquoi la mixité sociale est essentielle dans le domaine scolaire, tant elle permet de lutter contre les inégalités dès l’enfance. C’est tout l’enjeu du texte que nous examinons. La proposition de loi de Mme Colombe Brossel pose les bons diagnostics. collègue dresse le constat de la persistance de la ségrégation scolaire, malgré l’inscription de l’objectif de mixité dans la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Elle met également en lumière l’écart d’attractivité entre les établissements publics et ceux de l’enseignement privé sous contrat, qui accueillent une plus grande proportion d’élèves issus de milieux favorisés. Les outils dont disposent l’éducation nationale et les collectivités territoriales pour corriger ces tendances de fond ne manquent pas, puisque les collectivités territoriales peuvent, comme vous le savez, agir sur la sectorisation des élèves et la localisation des nouveaux établissements scolaires. La proposition de loi tend à actionner de nouveaux leviers en agissant par la contrainte. Elle vise, par exemple, à rendre obligatoire le partage d’un secteur de recrutement entre plusieurs collèges coexistant dans un périmètre rapproché. Elle étend par ailleurs la procédure Affelnet aux lycées privés sous contrat et conditionne leur financement public au respect d’une obligation de mixité sociale. Si nous sommes d’accord sur les constats, nous sommes en revanche en désaccord sur les solutions envisagées. Opposer établissements privés et établissements publics nous paraît d’autant moins pertinent que le secteur privé sous contrat participe déjà de manière importante à l’accueil des élèves boursiers. Ne faisons pas de l’enseignement privé, aux spécificités propres, un clone de l’enseignement public, au risque de gommer toute différence de nature entre eux. En outre, cela pourrait à terme légitimer le discours selon lequel plus rien ne justifie que cohabitent au sein de l’éducation nationale des établissements qui se ressemblent en tout point.

Vous ne tarderez pas à constater les effets notables de cette politique vertueuse en termes de progression des résultats, d’estime de soi, de cohésion scolaire et de respect mutuel auprès des enfants et adolescents. J’aimerais profiter de l’examen de cette proposition de loi pour rappeler l’existence d’un autre défi en matière d’égalité des chances, celui de la réussite des jeunes issus de la ruralité. En mars 2023, notre groupe soulignait, lors d’un débat, que la mixité sociale à l’école revêt une importance toute particulière en milieu rural. en milieu rural. Mon collègue Pierre Jean Verzelen indiquait qu’en milieu urbain, rural, dans les villes moyennes ou dans les métropoles, à chaque territoire correspond une boîte à outils en matière de politique de mixité sociale et scolaire. L’école républicaine doit en effet honorer ses promesses dans tous les territoires. Pour ces différentes raisons, la présente proposition de loi ne nous semble pas répondre de manière adaptée aux enjeux auxquels fait face l’éducation nationale ni aux fractures multiples qui divisent notre société. L’objectif de mixité sociale et scolaire doit être notre boussole durant les années à venir, au même titre que l’excellence et la laïcité. La méritocratie doit redevenir l’unique moteur pour tous les élèves de France. Je salue particulièrement les parcours d’excellence, qui font la fierté des élèves qui l’obtiennent et de leurs familles.

cette proposition de loi : oui, notre escalier social est en panne ; oui, il est indispensable de le reconstruire au plus vite. Pour le reste, nous retrouvons dans ce texte tous les marqueurs d’une gauche toujours plus encline à l’uniformisation et à l’étatisation. Pour quels résultats, mes chers collègues, sinon une crise inédite touchant tous les pans de l’éducation, dans laquelle s’enlise inexorablement notre système éducatif ?

alors qu’ont été éjectés tous les éléments de réussite scolaire – notes, appréciations, livrets, examens, bref, tous les outils de la méritocratie

de véritable boussole du pilotage de la répartition des élèves dans les établissements. En d’autres mots, les élèves ne seront plus perçus selon leur mérite, mais selon la seule détermination sociale. Voilà comment achever définitivement toute forme de méritocratie. Par ailleurs, alors que la Cour des comptes, rapport après rapport, invite à développer l’autonomie des établissements, vous proposez au contraire une méthode verticale, contraignante en fixant de rigides barrières, qui seront de toute façon contournées en ce qu’elles tournent le dos aux réalités de la vie quotidienne.

Je crois davantage à une école qui pratique la différenciation dans les territoires aux besoins éducatifs particuliers, qui envoie ses meilleurs professeurs là où ils sont indispensables, qui repense son rapport aux territoires en partenariat avec les collectivités, qui revoit sa carte de l’éducation prioritaire et dessine une nouvelle politique de la grande ruralité. Une autre lubie chère à la gauche innerve également ce texte : celle qui vise, au nom de la mixité scolaire et sociale, à remettre méthodiquement en cause les fondements de la liberté de l’enseignement. Purgeons en premier lieu une caricature : beaucoup d’établissements privés sous contrat participent à l’effort de mixité sociale et scolaire. Toutefois, il est vrai que l’enseignement privé sous contrat

à la méritocratie républicaine ? Il ne cesse de démontrer, dans sa grande diversité, qu’insuffler de la souplesse et de la liberté dans l’organisation pédagogique

aucune planification, aucune uniformisation, aucune idéologie centralisatrice ne permettront de reconstruire l’escalier social. Seul le pourra un grand vent de liberté et d’autonomie, que j’appelle de mes vœux. Pour cette raison, le le groupe Les Républicains votera résolument contre cette proposition de loi, qui, loin de présenter des solutions pour la mixité sociale, n’a d’autre objet que de conforter un dogmatisme qui mine depuis trop longtemps l’école de la République. Quelle

inégalités naturelles, inégalités de dons ». Très bien ! Si, depuis, les politiques publiques ont heureusement pris en considération cette problématique, la France reste malgré tout l’un des pays de l’OCDE où les déterminismes sociaux pèsent le plus sur la réussite scolaire des élèves. De fait, il est souvent démontré qu’un manque de mixité scolaire nuit à la réussite de tous les élèves et à la promesse d’égalité des chances de l’école républicaine.

contre 106 pour les collèges publics hors éducation prioritaire. Dans ce contexte, sous l’égide des gouvernements successifs depuis 2017, l’ensemble des acteurs ont été mobilisés afin de réduire la ségrégation sociale des établissements scolaires publics de 20 % d’ici à 2027.

géographiquement, qui disposent d’IPS différents. Des réflexions ont commencé à être menées afin de renforcer la mixité sociale au sein de ces mêmes

De plus, afin d’accompagner et d’inciter les familles les plus modestes à inscrire leurs enfants dans les internats d’excellence, la prime d’internat a été revalorisée. Les efforts entrepris sont donc réels. Ils portent déjà leurs fruits, comme en témoigne la note du conseil scientifique de l’éducation nationale d’avril 2023. Il est établi que le renforcement de la mixité sociale n’a pas entraîné d’évolution significative, positive ou négative, des résultats scolaires à l’échelle des établissements concernés. En revanche, ceux des élèves les plus défavorisés qui sont scolarisés dans un établissement socialement plus favorisé ont vu leurs résultats scolaires progresser. De plus, contrairement à ce que certains pouvaient craindre, l’amélioration de la mixité scolaire et sociale n’a pas entraîné une mobilité massive vers l’enseignement privé sous

tacite qui existe à la fois avec les établissements privés, mais également avec les parents d’élèves, qui disposent de la liberté de choisir le type d’école dans lequel ils souhaitent scolariser leurs enfants. Au lieu de contraindre les parents en ravivant la guerre scolaire au nom de la mixité sociale, nous préférons faire preuve de pédagogie et accompagner l’ensemble des acteurs vers une plus grande mixité sociale dans nos écoles.

la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. Et la réponse se trouve dans l’école, dans l’orientation ». Ces mots sont ceux prononcés par Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux Français pour l’année 2023. Dix ans plus tôt, en 2013, la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République assignait au service public de l’éducation la mission de veiller à « la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Dix années plus tard, l’objectif est loin d’être atteint. Rappelons les chiffres : l’enseignement privé compte 40 % d’élèves d’origine sociale très aisée, contre 20 % dans le public. À l’inverse, 42 % des élèves du public sont issus de milieux sociaux défavorisés, contre 18 % dans le privé. En ce qui concerne les collèges, si la ségrégation sociale au sein des établissements tant publics que privés tend à diminuer, les disparités

l’éducation nationale a signé avec l’enseignement catholique un protocole d’accord afin de renforcer les mixités sociale et scolaire. Par ce texte, l’enseignement privé sous contrat s’engage, de manière non contraignante, à augmenter la part de ses élèves boursiers. Si cette démarche est positive pour la mixité sociale, elle n’a pas vocation à favoriser la mixité scolaire. En effet, elle peut conduire à sélectionner les élèves boursiers ayant les meilleurs résultats et à priver ainsi le public de ses meilleurs élèves, alors que ce dernier doit déjà plus souvent faire face à des handicaps sociaux. Il faut aussi citer les filières d’excellence, qui peuvent mener à une ségrégation scolaire au sein d’un même établissement : je pense, par exemple, à la section européenne, à la section orientale ou encore à l’apprentissage des langues anciennes. les lycées, l’intégration des lycées Louis le Grand et Henri IV dans le système d’affectation Affelnet a eu des résultats prometteurs. Elle a permis de diversifier les profils des élèves admis, d’un point de vue tant social que scolaire.

À quoi bon calculer un IPS pour ne pas le diffuser ? L’IPS permet de repérer les inégalités : utilisons le comme outil d’harmonisation. À ce sujet, le groupe RDSE présentera un amendement visant à faire de l’IPS un critère dans le calcul des contributions communales aux dépenses de fonctionnement des classes : plus l’IPS est faible, plus les dépenses seront élevées, et inversement.

En 2023, l’ancien ministre de l’éducation nationale, M. Pap Ndiaye, a annoncé un objectif de « réduction de la ségrégation sociale » des établissements scolaires publics de l’ordre de 20 % d’ici à 2027. Des mesures ont été prises en ce sens : directives, ouverture de sections internationales et de classes à horaires aménagés, valorisation de l’internat d’excellence… À l’échelle l’échelle locale, les collectivités territoriales disposent de plusieurs outils pour favoriser la mixité sociale. Les résultats des premières expérimentations sont d’ailleurs encourageants.

Tout d’abord, l’instauration d’un impératif de mixité sociale et scolaire n’est pas en phase avec le besoin de simplification et d’autonomie des collectivités locales. ces dernières étouffent sous le contingent de normes et de contraintes à respecter, il ne semble pas judicieux d’ajouter des obligations supplémentaires. Par ailleurs, la généralisation d’outils peut être intéressante, mais veillons à ne pas tomber dans une centralisation contre productive.

dont j’ai pu faire mention dans de précédentes interventions : un élève du privé sous contrat coûte en moyenne à l’État 60 % du coût d’un élève dans le public… En conditionnant le financement de l’enseignement privé, cette proposition de loi remet en cause les principes de la loi Debré. Interrogeons nous plutôt sur le fond du problème. Le chef d’un établissement privé sous contrat vendéen me faisait récemment part de son désarroi : en un an, près d’une dizaine de familles ont dû retirer leurs enfants de son établissement, faute de pouvoir subvenir à l’ensemble des frais afférents à leur scolarité.

euros dans le public. En d’autres termes, il s’agit non pas tant d’imposer plus de mixité sociale aux établissements privés sous contrat que de se demander comment permettre aux familles de tous horizons de financer la scolarisation de leurs enfants dans le privé.

Je tiens toutefois à saluer la démarche de l’auteure et le travail de la rapporteure, qui nous permettent de débattre d’une thématique importante. Les nombreux travaux de la commission illustrent la nécessité d’avancer sur les questions d’éducation. de pause méridienne, dite loi Vial, mais aussi aux conclusions de la mission d’information sur les modalités de formation des enseignants, que j’ai menée avec Max Brisson. Brique après brique, nous devons consolider les fondations de l’école de demain. Cette construction ne peut se faire que sur le temps long. Pourtant, en une année, l’éducation nationale a accueilli pas moins de quatre ministres. Une telle valse au sommet du premier budget de l’État rend impossible le développement de politiques publiques volontaires et pérennes. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie vivement Mme Colombe Brossel et ses collègues du groupe socialiste de nous permettre de confronter nos conceptions politiques sur le rôle et les obligations de l’enseignement catholique dans notre République laïque du XXI siècle. Il serait vain de débattre de son financement sans s’interroger préalablement sur le cadre juridique dans lequel il évolue. Lors de son audition par notre commission, M. Philippe Delorme, secrétaire général de l’enseignement catholique, nous a dit que les établissements qu’il représente assurent une mission de service public. Certains d’entre vous, mes chers collègues, ont considéré avec lui que l’enseignement catholique était l’une des composantes du service public de l’éducation nationale. Pourtant, l’enseignement catholique ne le revendique pas. Son statut, adopté par la Conférence des évêques de France le 18 avril 2013, précise qu’il se place « dans une logique de contribution au service éducatif de la Nation », mais que « le caractère ecclésial de l’école est inscrit au cœur même de son identité d’institution scolaire Cette volonté de dispenser à tous les élèves et dans toutes les matières un enseignement fondé sur l’Évangile distingue radicalement l’école confessionnelle de l’école publique laïque, dont la mission est de délivrer des connaissances fondées sur la liberté de pensée, la libre recherche, les progrès de la raison et de la science, et donc libérées de tout dogme et de toute croyance, pour reprendre la définition qu’en donnait Condorcet en 1792. Le code de l’éducation, en son article L. 442 5, conditionne la conclusion d’un contrat d’association avec l’État à « la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public M. Jean François Canteneur, directeur diocésain de l’enseignement catholique de Paris, souligne cette aporie et déclare : « Il Il va falloir dialoguer sur la notion de laïcité dans l’enseignement catholique. Aujourd’hui, l’État n’a pas la compétence pour juger de la qualité d’un enseignement religieux. Cette revendication pose le problème de la nature de ce « caractère propre » que la loi reconnaît aux établissements sous contrat. Se rapporte t il à la totalité des enseignements qu’ils dispensent ou seulement à la catéchèse ? termes, le financement de l’État et des collectivités doit il se limiter aux seules matières du programme national ? La question est financière, mais aussi juridique, car une majorité des parents qui confient leurs enfants à ces écoles ne le font plus pour des raisons religieuses. comment est il possible de donner un enseignement catholique à des élèves qui ne le sont pas et avec des professeurs qui ne le sont plus, tout en respectant la liberté de conscience des uns et des autres ?

Pis, certains de leurs dirigeants assument totalement de recruter en priorité les enfants des familles les plus riches. Ainsi le directeur diocésain de l’enseignement catholique de Paris déclare t il : « Plus on dira que l’école privée est une école de l’entre soi, de gens privilégiés, plus elle attirera. On ne peut se réjouir de cela, mais c’est ainsi. » Madame la ministre, comment pouvez vous accepter que l’argent de l’État,

aux objectifs de mixité qui ont été fixés à maintes reprises dans les précédentes lois ou précédents protocoles, le dernier datant seulement de 2023. En cherchant à assurer la mixité sociale et scolaire, ce texte pointe largement l’enseignement privé. Si le sujet est bien plus large, quelques précisions s’imposent.

que l’indice de position sociale et la procédure Affelnet concernent tous les établissements. À ce stade, ils ne doivent pas se transformer en instruments de chantage idéologique, ainsi que pourrait le laisser entendre l’article 1, en y conditionnant les ouvertures de classe ou le versement des financements.

que certains établissements privés assurent une mission de service public en perdurant dans des déserts académiques, là où l’État ne parvient plus à maintenir des classes. L’interdiction d’ouverture ne peut que provoquer une chute collective dans des zones sous dotées.

aux particularités locales. Il serait plus judicieux de donner à tous les établissements les moyens – pas seulement financiers – de se doter de ces deux qualités. Cette agilité, qui ne peut être régie par des circulaires nationales, permettrait le retour de l’autorité et une souplesse pédagogique. Dans ce pays, où la norme devient reine, il nous semble également indispensable de laisser aux familles le libre choix de la scolarisation de leurs enfants ; il faut les inciter à oser, comme vous l’avez souligné, madame la ministre. L’urgence de la situation éducative du pays, à tous les degrés, nous appelle

permettez moi de vous rappeler l’article 60 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privé liés à l’État par contrat, dans un délai d’un an à

Merci

Mme la rapporteure.

évoqué l’argent de l’État, je parlerai de celui des régions. La seule région Auvergne Rhône Alpes, présidée entre 2016 et 2024 par Laurent Wauquiez, a augmenté de plus de 266 % les aides facultatives accordées aux lycées privés. Cela représente 260 millions d’euros

Vous nous avez dit que vous ne seriez pas la ministre du tri social, mais vous laissez faire le mouvement, voire vous l’encouragez en vantant le si décrié et par ailleurs peu mis en œuvre « choc des savoirs

pour cette si belle école de la République, La République française est laïque et sociale et je pense que les écoles privées ne sont ni laïques ni sociales. C’est un peu court ! Certaines d’entre elles, toujours plus nombreuses malheureusement, ont décidé de sélectionner leurs élèves, en retenant des enfants issus des classes sociales supérieures. Est ce un choix qui est conforme à leur pastorale ? C’est à leurs responsables d’en juger en conscience. Pour nous, il est inadmissible que ces établissements continuent de recevoir la manne publique, alors qu’ils entretiennent le séparatisme scolaire. Vous nous avez donné une information capitale, madame la ministre, et je pense que c’est un éclaircissement fondamental, sur le « caractère propre » des établissements privés. Vous nous avez dit que le financement de l’État ne portait que sur l’enseignement des programmes nationaux, c’est à dire la partie nationale et laïque

pour adapter les outils aux publics auxquels ils sont confrontés. Je rappellerai enfin que la majorité sénatoriale a été force de proposition

sur les travées de la majorité sénatoriale – elles n’étaient pas très fournies, je peux vous l’accorder –, d’une parole rare, mais cela ne veut pas dire qu’il y avait approbation. Les votes l’ont montré. Madame la ministre, c’est la première fois que vous travaillez avec nous dans cette assemblée, je tiens à vous assurer que, même sur le sujet de l’école, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport